prises pour son application, la commission des finances a émis un avis favorable- 18 voix pour, aucune voix contre et 3 bulletins blancs -à la nomination de M. Robert Ophèle aux fonctions de président de l'Autorité des marchés financiers. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs au sein de deux organismes extraparlementaires. La commission de la culture a proposé les candidatures de M. Jean-Pierre Leleux et de Mme Françoise Férat pour siéger au sein de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, et de M. Christian Manable pour la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Ces candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure. Le Conseil

Sénat. L'ordre du jour appelle l'examen de six projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces six projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Secrétariat de l'accord relatif

autorisant la ratification du traité entre la République française et la République tchèque relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (projet n° 338, texte de la commission n°

et la République portugaise relatif à l'assistance et à la coopération dans le domaine de la sécurité civile et l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à l'assistance et à la coopération dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles

l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs,

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant création de l'établissement public Paris La Défense que nous allons examiner a été déposé devant le Parlement le 10 mai 2017

relevant du domaine de la loi ayant pour objet : la création d'un établissement public local associant l'État, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour l'aménagement, la gestion et la promotion du territoire de " Paris La Défense " ; la définition des pouvoirs spécifiques attribués à l'État ; la définition du périmètre d'intervention géographique de cet établissement, en concertation avec les communes concernées ; la substitution de cet établissement à l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense et à l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche ». Cela n'a rien de simple depuis longtemps En effet, le modèle de gestion et de développement du quartier d'affaires de La Défense, reposant sur deux établissements- l'un compétent en matière d'aménagement, l'autre en matière de gestion -, ne répond pas aux enjeux de développement et de rayonnement auxquels le quartier C'est pourquoi le précédent gouvernement- comme vous le savez, il y a une continuité de l'État -a engagé un processus de réunion de l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, l'EPADESA, et de l'établissement public de gestion de La Défense, dénommé Defacto, afin de renforcer son modèle économique et mieux associer les collectivités dans sa gouvernance. L'ordonnance déposée sur le bureau des assemblées le 4 mai dernier prévoit ainsi la création, au 1 janvier 2018, d'un établissement public local se substituant aux deux établissements. La décentralisation de cet établissement confie pleinement la responsabilité du développement de La Défense aux collectivités territoriales, notamment au département des Hauts-de-Seine, qui sera majoritaire au conseil d'administration, ce que tout le monde a bien entendu. Les communes de Courbevoie, Nanterre, Paris et Puteaux, ainsi que la région d'Île-de-France et la métropole du Grand Paris seront également représentées. Par l'intermédiaire du préfet de région, l'État restera présent au sein de l'établissement, dans le but de veiller au bon fonctionnement des services publics dont l'établissement aura la charge. La commission a souhaité revenir sur ce rôle. Je présenterai un amendement visant à rétablir les missions de contrôle du préfet, dans un souci de coordination de l'action de l'État sur le territoire de La Défense et de celle de l'établissement.

et des opérations nécessaires au bon fonctionnement des services publics, notamment celles qui sont assurées par la RATP, SNCF réseau, la SNCF ou la la SGP. S'agissant du patrimoine de l'établissement, l'ordonnance qu'il est question ici de ratifier prévoit que les droits, biens, obligations et personnels de l'EPADESA et de Defacto seront transférés à titre gratuit. Toutefois, les parcs de stationnement appartenant à l'EPADESA feront retour à l'État et seront mis à disposition du nouvel établissement pour une durée de soixante Je sais sur ce point qu'un bon nombre d'entre vous, mesdames, messieurs les parlementaires, a souhaité revoir le texte et prévoir le transfert des parcs de stationnement de l'EPADESA dans les mêmes conditions que les autres biens des établissements fusionnés. me semble-t-il, sur les équilibres construits au cours des derniers mois entre le Gouvernement et les élus de ce territoire. Le Gouvernement souhaite préserver les équilibres de l'ordonnance, qui sont le résultat de longues discussions de longues discussions entre l'État et le département. Il ne s'agit pas d'être fermé aux propositions du Parlement. Vous savez qu'à titre personnel, j'attacherai toujours la plus grande importance à ce que proposent les parlementaires

En effet, le nouvel établissement public Paris La Défense exercera une compétence d'aménagement sur un périmètre comprenant tout ou partie du territoire correspondant à celui des opérations d'intérêt de l'actuel EPADESA et couvrant une partie des communes de Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre et Puteaux. Ce périmètre sera délimité par décret en Conseil d'État pris après avis des communes précitées. Il exercera également une compétence de gestion sur un périmètre comprenant tout ou partie du territoire correspondant à celui de l'opération d'intérêt national correspondant à l'actuel périmètre d'intervention de Defacto et couvrant une partie des communes de Courbevoie et Puteaux. Ce périmètre sera délimité par décret en Conseil d'État pris après avis de ces deux communes. Enfin, un périmètre de compétence exclusive de l'établissement est établi, qui correspond aux deux périmètres d'opération d'intérêt national. Sur ce point, ce point, la commission a souhaité élargir l'assiette potentielle du périmètre d'intervention de Paris La Défense en matière d'aménagement au-delà du périmètre que je viens de citer, en supprimant l'avis de ces communes préalable au décret en Conseil d'État fixant les périmètres d'intervention de l'établissement respectivement prévus à ces mêmes articles, en le remplaçant par une concertation. Je proposerai à la Haute Assemblée un amendement visant revenir à la rédaction antérieure quant au périmètre d'intervention. En ce qui concerne les modalités de concertation des communes, je vous proposerai d'ajouter à l'avis proposé par le Gouvernement la notion de concertation introduite par la commission. un des enjeux majeurs de cette fusion est de permettre un financement équilibré des travaux d'entretien et de mise aux normes de l'ensemble des biens et espaces publics situés dans le périmètre de gestion de l'établissement, dont la vétusté, il faut le reconnaître, nuit aujourd'hui à La Défense, à son fonctionnement et, aussi, à son image, ce qui est particulièrement important s'agissant d'un quartier dont le fonctionnement est tout à fait primordial pour l'image, d'ailleurs, du territoire tout entier. Les collectivités devront donc apporter une contribution financière couvrant le reste à charge à financer en matière de gestion un document d'engagement négocié. Ces engagements, pris sur dix ans, permettront de décliner les objectifs, la stratégie et les moyens qui seront mis en oeuvre par l'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements, pour réaliser 360 millions d'euros d'investissements sur dix ans pour la remise en état des biens et ouvrages publics dans le quartier d'affaires, d'annoncer à l'occasion de la Conférence nationale des territoires une conférence territoriale du Grand Paris. Cet outil décentralisé devra contribuer à renforcer la place de La Défense dans la compétition internationale entre les grands centres d'affaires. Vous l'avez compris, et cela a été l'objet de très longues discussions qui ont eu lieu depuis longtemps, il s'agit de sortir d'une situation compliquée, trop compliquée, de prendre en compte la réalité de la situation d'entretien de l'ensemble de ce quartier et d'essayer de trouver, dans le meilleur consensus possible, les moyens de remédier à ces difficultés de fonctionnement, à ces retards d'entretien, pour redonner à ce quartier, extrêmement important pour l'image de toute l'Île-de-France, les moyens d'être à la hauteur

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission, mes chers collègues,

ardent défenseur des territoires. L'heure du Brexit se rapproche, et de nombreuses activités basées à Londres, qu'il s'agisse de certaines agences européennes- notamment l'Autorité bancaire -ou des entreprises du secteur de la finance, vont devoir réinstaller leur activité sur le continent, dans un État membre de l'Union. Ces entités auront besoin de volumes de bureaux très importants, dans un environnement favorable aux services, desservi par les infrastructures nécessaires où elles retrouveront un écosystème familier, à proximité de leurs interlocuteurs. Où iront-elles ? À Francfort ? Milan ? Bruxelles ? Ou bien, et ce serait fort naturel, en France ? ? Ce lieu idéal existe effectivement déjà dans l'Hexagone : il s'agit de La Défense, le premier quartier d'affaires européen par l'étendue de son parc de bureaux. Celui-ci regroupe environ 2 950 entreprises, dont 14 des 20 premières entreprises nationales et 15 des 50 premières entreprises mondiales. 180 000 salariés qui y travaillent chaque jour et 245 000 mètres carrés de commerces permettent d'accueillir les activités les plus diverses. La gouvernance du quartier de La Défense est, depuis le décret le 9 septembre 1958, du ressort de l'Établissement public pour l'aménagement de la région de La Défense, l'EPAD, qui se trouve être un établissement public à caractère industriel et commercial, dont la mission est d'aménager le site pour le compte de l'État et des collectivités locales concernées. Toutefois, on observe que, depuis soixante ans, les pouvoirs publics n'ont jamais su trouver une gouvernance adaptée et un financement pérenne. L'EPAD a connu de nombreuses évolutions institutionnelles, qui ont notamment abouti à la création de l'Établissement public de gestion de La Défense, devenu Defacto en 2010, soulageant l'EPAD de sa mission d'exploitation des espaces publics dont il s'acquittait par défaut. Prise sur le fondement d'une habilitation consentie par l'article 55 de la loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, l'ordonnance du 3 mai 2017 portant création, à compter du 1 janvier 2018, 2017 portant création, à compter du 1 janvier 2018, de l'établissement public Paris La Défense constitue une première réponse institutionnelle à ces enjeux et l'aboutissement d'une réflexion engagée par l'État en concertation avec les acteurs concernés, singulièrement les collectivités territoriales, depuis mai 2016. Le projet de loi qui vous est soumis a donc pour objet de la ratifier. Dans le cadre de la loi relative au statut de Paris, le Parlement a donc habilité le Gouvernement à créer, par ordonnance, un établissement public unique se substituant à Defacto et à l'EPADESA, compétent à la fois pour l'aménagement, la gestion et la promotion du quartier d'affaires de La Défense. Cette habilitation prévoyait un pilotage unifié et un financement solide du quartier d'affaires, en vue de pérenniser son attractivité. L'ordonnance entrera en vigueur et le nouvel établissement public sera créé le 1 janvier 2018. Si la commission des lois souscrit à la plupart des dispositions contenues dans l'ordonnance, elle constate que plusieurs d'entre elles excèdent le périmètre de l'habilitation ou sont contraires aux objectifs initiaux voulus par le législateur, en particulier en matière de simplification et d'efficacité du nouvel établissement public local. Voilà pourquoi elle a adopté sept amendements qui pourront rétablir cette volonté exprimée par le législateur, même si nous entendons bien les arguments qu'a invoqués à l'instant M. le ministre. Ainsi, sur la question des périmètres d'intervention strictement délimités, la commission a considéré qu'ils étaient peu susceptibles d'évolution et en a supprimé les limites prévues. Cela permettra de redessiner, si besoin, les périmètres d'intervention du nouvel établissement public local après concertation avec les communes concernées- plutôt qu'après un simple avis -, afin d'actualiser les périmètres de La Défense, au lieu de se contenter de reprendre le coeur historique du quartier d'affaires au moment du Brexit, dont j'évoquais les opportunités. Pour conférer à l'établissement public davantage de souplesse, la commission a également inscrit dans le texte de l'ordonnance l'autorisation explicite de créer des filiales, d'acquérir ou de céder des participations dans des sociétés publiques locales, groupements ou organismes, y compris des sociétés publiques locales d'aménagement, dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions par Paris La Défense. Elle a supprimé le pouvoir donné au préfet de Région de suspendre le caractère exécutoire des décisions du conseil d'administration de Paris La Défense pour atteinte au bon fonctionnement des services publics. En effet, elle a considéré que les pouvoirs spécifiques de l'État à l'égard des décisions du nouvel établissement public étaient susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement des services publics et semblaient méconnaître les compétences dévolues à Paris La Défense en matière de gestion des services d'intérêt général dans son périmètre d'intervention. Enfin, la commission a supprimé, à l'article 3 de l'ordonnance, sous réserve d'éléments complémentaires fournis par les représentants de l'État, la disposition excluant les parcs de stationnement du transfert en pleine propriété des biens de l'EPADESA vers le nouvel établissement Paris La Défense. Telles sont donc les améliorations qu'a souhaité apporter la commission au projet de loi de ratification et qu'elle vous propose d'adopter en ces termes. Mes chers collègues, monsieur le ministre, le Brexit est une chance pour notre économie et constituerait une opportunité historique pour le quartier de La Défense, qui renforcerait sa place européenne et internationale. Figure emblématique trônant au milieu d'une forêt de gratte-ciel et de leur architecture qui parle au futur, se trouve la Grande Arche. Tête de pont de cette perspective qui court jusqu'au Louvre en passant par l'Arc de Triomphe et la Concorde, l'Arche de la Défense est une porte d'entrée qui ne demande qu'à s'ouvrir sur les projets de ceux qui pensent que l'avenir est une chance plutôt qu'un risque. C'est la raison pour laquelle il faut que la gouvernance de La Défense soit à la mesure de l'enjeu et qu'elle soit pensée, dessinée et mise en oeuvre comme l'outil qui l'aidera à relever ce fantastique défi. La parole est à M.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la vice-présidente de la commission, mes chers collègues, l'ordonnance qui nous est soumise aujourd'hui pour ratification me semble intervenir trop tard ou trop tôt. trop tôt. Trop tard, parce que depuis 2011, date de mon arrivée au Sénat, je milite avec d'autres collègues et élus des Hauts-de-Seine pour que la gestion du quartier d'affaires de La Défense puisse s'opérer dans un réel partenariat entre l'État et les collectivités locales, tout en y associant les habitants qui y vivent, les salariés qui y travaillent et les entreprises qui y créent des activités. Nous pensons depuis longtemps que la cogestion de ce quartier entre deux établissements publics-

Nous pensions qu'un établissement unique permettrait une meilleure gestion à moyen et long terme, et qu'une réelle ouverture de fonctionnement éviterait l'entre soi et certaines dérives dans la gouvernance. dérives dans la gouvernance. Nous continuons de penser que la création de cet établissement devrait se faire en toute transparence lors d'une conférence qui réunirait l'ensemble des acteurs impliqués dans ce quartier, c'est-à-dire les maires, les élus municipaux des villes de Courbevoie, de La Garenne-Colombes, de Paris, de Nanterre, de Puteaux, les élus régionaux et départementaux, mais aussi les parlementaires et les représentants de l'État. Pourquoi Paris ? Paris ne En effet, en novembre 2016, dans le projet de loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, nous avons découvert non sans étonnement l'article 38, qui portait sur la création, par voie d'ordonnance, d'un établissement unique pour gérer ce quartier d'affaires. Seulement, cette proposition de création a été faite en catimini, en se basant sur un rapport commandé par le Premier ministre de l'époque, M. Manuel Valls, processus a duré des mois ! Ce document, je n'ai, en tant que parlementaire du département, jamais pu en avoir connaissance ! Encore aujourd'hui, monsieur le ministre, après l'avoir réclamé à votre prédécesseur,

! Ce texte arrive peut-être un peu tardivement, parce que pendant cinq ans les problèmes relatifs à la mise à niveau des équipements publics de ce quartier, l'entretien de la dalle, des tunnels qui commencent à être atteints par l'usure propre à ce type d'installation, n'ont pas été traités et que les dégradations n'ont pas cessé de progresser.

trop tôt ... Trop tôt, mes chers collègues, parce qu'entre 2011 et aujourd'hui, est née, en 2016, la métropole du Grand Paris. Il faudra encore du temps pour que cette dernière prenne toute son ampleur. Du temps, et aussi une volonté politique claire. Il faut l'avouer, la clarté n'a pas présidé à sa création, la loi

le discours qu'il a prononcé lundi dernier, lors de la Conférence nationale des territoires qui s'est tenue au Sénat. Permettez-moi de le citer : « Si nous voulons que le Grand Paris réussisse à l'échelle de ce qu'est la compétition internationale, si nous voulons produire la richesse pouvoir la répartir harmonieusement sur le territoire, nous avons besoin de simplifier drastiquement les structures. » Et il complète ses propos en indiquant qu'il va réunir cet automne une conférence territoriale du Grand Paris, « qui devra se refonder autour d'un projet ambitieux de développement de la première métropole française, au sein de la région capitale, et aboutir à une organisation institutionnelle stabilisée et efficace ». À l'automne, le fonctionnement institutionnel de la métropole du Grand Paris va donc être discuté, renforcé, mais d'avance, on a le sentiment qu'on lui soustrait, cette ordonnance, une possibilité de peser économiquement, car on lui retire la gestion du quartier d'affaires de La Défense pour la confier au département des Hauts-de-Seine. On peut s'interroger sur la stratégie globale qui préside à ces décisions. Ce texte arrive donc peut-être un peu trop tôt. Trop tôt pour être en cohérence avec les projets présidentiels et pour tenir compte des perspectives de développement

consacrée presque exclusivement au seul quartier d'affaires de ce département ? Sur quelles aides pourront compter les autres secteurs d'activité des Hauts-de-Seine, notamment le port de Gennevilliers, le centre économique d'Issy-Boulogne ou encore celui d'Antonypole ?

Ensuite, cette ordonnance recèle deux questions juridiques constituant en réalité deux anomalies démocratiques. Le 30 juin dernier, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a désigné par anticipation ses neuf représentants au conseil d'administration du futur établissement sans tenir compte des délais d'application fixés par l'ordonnance et par son décret d'application, qui prescrivent, précisément, que cette démarche doit être faite après le 1 janvier 2018, et non six mois avant. Monsieur le ministre, que vaut cette désignation préalable ? D'autant plus que, parmi les neuf personnes désignées, aucune ne représente l'opposition au sein du conseil départemental. Je ne voudrais pas être polémique, mais je dirai simplement qu'il nous appartient à nous, législateurs, de corriger ce comportement que je juge peu peu respectueux des usages et des bonnes pratiques démocratiques, en rappelant l'importance du pluralisme des opinions politiques dans la représentation des élus au sein de ces instances. En conclusion,

Monsieur le président, monsieur le ministre- je vous adresse mon amical salut-, mes chers collègues, le projet de loi qui nous occupe aujourd'hui, qui vise à la création, par fusion de l'EPADESA et de et de Defacto, d'un établissement public unique nommé Paris-La Défense, revêt des enjeux politiques et financiers colossaux. Il serait hypocrite de le cacher. Les intentions affichées par certains d'en faire, bien au-delà du quartier d'affaires historique, le réceptacle des retombées possibles du Brexit le prouve. Je ne reviendrai pas sur l'historique des séparations et fusions successives qui jalonnent ce dossier et des querelles qu'il a occasionnées. Mon groupe, l'année dernière, s'était prononcé favorablement sur l'article 55 de la loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain approuvant la création d'un établissement public local unique. Nous avions d'ailleurs défendu des amendements visant à clarifier le périmètre et à réagir à l'introduction en dernière minute, par amendement du gouvernement, du conseil départemental dans la liste des acteurs associés au sein de cet établissement public local. Aujourd'hui, nous franchissons une étape de plus avec la ratification de l'ordonnance portant création de cet établissement public. Je voudrais dire un mot d'abord sur les personnels de ces deux établissements. L'ordonnance, ainsi que nos précédents débats, est quasi muette à leur sujet, si ce n'est pour dire qu'ils seront transférés au nouvel EPL au même titre que les « biens, droits et obligations » J'attire votre attention, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur leurs vives inquiétudes, du fait de multiples interrogations laissées sans aucune réponse. En l'état, le texte issu des travaux de la commission des lois ne nous satisfait pas. Notre vote final dépendra donc du sort qui sera réservé à nos amendements, notamment nos amendements nos 1 et 2 rectifié . Le premier point de divergence avec la commission et M. le rapporteur porte sur le périmètre. Vous proposez de supprimer toute notion de « périmètre », allant ainsi à l'encontre des engagements du Premier ministre de l'époque, de la ministre du logement devant les deux assemblées et de la rédaction même de l'article 55, autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Cela questionne à nouveau sur le recours à l'ordonnance pour légiférer sur cette question. Pour justifier la réécriture de l'article 2 de l'ordonnance, vous nous expliquez, monsieur le rapporteur, que la définition de ces périmètres fera l'objet de « décrets en Conseil d'État pris après avis des communes concernées et au plus tard dans les six mois suivant la création de cet établissement public local, soit le 1 juillet 2018 ». Soyons précis : les décrets pourront intervenir après la création de l'EPL. On créerait ainsi l'EPL sans avoir au préalable défini son périmètre, soit son ADN. Étrange méthode Ce n'était pas l'intention du législateur au moment de voter l'article 55 du projet de loi dont vous étiez déjà le rapporteur, monsieur Darnaud, et c'est bien pour cela qu'un périmètre avait été déjà délimité.

toutes les opérations se fassent une convention conclue entre le territoire concerné et l'EPL. C'est d'ailleurs parfaitement conforme à la pratique qui a cours entre l'EPADESA et les communes, comme nous l'ont rappelé les représentants au comité d'entreprise des salariés de l'EPADESA, que nous avons, nous, auditionnés. Notre proposition de rédaction ne sort donc pas de nulle part. Elle est cohérente avec ce qui se pratique déjà sur le terrain. Il n'est donc pas vrai de dire que nous proposons juste un retour un retour à la rédaction initiale. Nous formulons d'autres propositions d'amendements ayant notamment pour objet la composition du conseil d'administration. Nos craintes, exprimées en décembre dernier, quant à l'introduction du conseil départemental dans la liste des acteurs associés, se confirment à la lecture de la composition des membres désignés par ce même conseil. Nous proposons donc d'introduire un peu de « pluralisme », et donc d'équilibre, dans la composition du conseil d'administration. Ce sera l'objet de l'amendement n° 2 et de son sous-amendement. J'ai parlé « d'équilibre Je crois que c'est vers quoi nous devons tendre, s'agissant de ce territoire qui accueille certes un quartier d'affaires avec ses salariés, mais aussi des habitants, des services publics, des activités. Ne refaisons pas l'erreur de ne prendre en compte que le seul prisme économique, financier devrais-je dire, car les enjeux en termes d'équipements, de logements, notamment sociaux, de services publics et de défi environnemental, et au final de « vivre ensemble », sont considérables. Ce projet, au sein d'un département certes riche, mais inégalitaire et en proie à de fortes disparités, peut permettre de rééquilibrer la balance en faveur des populations et des territoires. Je souhaite donc,

le Président de la République a décidé que la simplification des structures du Grand Paris se fera dès cet automne après la tenue de la conférence territoriale du Grand Paris. L'enjeu est crucial pour la France. Il s'agit de « produire la richesse qui pourra être ensuite répartie harmonieusement sur le territoire À mon sens, la consolidation de l'attrait de la région capitale va de pair avec le projet de rénovation du développement économique du quartier d'affaires porté par l'ordonnance créant l'établissement public Paris La Défense. En effet, Paris La Défense est un axe majeur du développement du Grand Paris. Il constituera l'un de ses principaux moteurs économiques, et l'un des symboles de son dynamisme international. Face aux trop nombreuses difficultés qui ont nui à l'attractivité de La Défense depuis les années 2000, cette ordonnance doit permettre de trouver un financement durable et une gouvernance stabilisée pour les années à venir. Il s'agit notamment de constituer une unité de pilotage en remédiant à la décision prise en 2007 de séparer les fonctions d'aménagement et de gestion confiées à deux établissements distincts, décision qui avait créé une confusion des responsabilités et gêné le développement du quartier d'affaires. L'inéquitable répartition de la charge financière entre l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche et Defacto avait conduit à repousser les travaux depuis de trop nombreuses années, compromettant le fonctionnement quotidien du quartier. La mise aux normes de sécurité des tunnels et sous-sols, la répartition des réseaux d'assainissement, le désamiantage sont autant d'investissements indispensables que l'établissement public devra désormais mener de front sur une dizaine d'années, pour un montant minimum estimé à 360 millions d'euros. La Cour des comptes a alerté pendant longtemps sur le manque de vision commune concernant l'avenir du quartier de La Défense. Des interrogations demeurent aujourd'hui à ce sujet. Il serait nécessaire de connaître au plus vite, d'une part, les modalités de la participation financière renforcée des collectivités, participation requise pour accompagner un programme d'investissement pluriannuel, et, d'autre part, les orientations stratégiques du nouvel établissement,

La décentralisation de l'établissement, près de soixante ans après sa création, permet enfin de confier la responsabilité de son développement et de son entretien aux collectivités territoriales concernées, marquant ainsi une nouvelle étape de l'aménagement du Grand Paris. Quant à l'État, il ne se dégage pas totalement. Il siégera au conseil d'administration de la nouvelle structure aux côtés des représentants des collectivités locales, avec un objectif de cohésion, d'efficacité et de réalisme. Avec cette décentralisation, les communes gagnent en pouvoir sur le choix des projets puisque les droits de vote au sein du conseil d'admiration sont conditionnés par la participation financière des collectivités, encore que j'ai entendu la remarque de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen indiquant qu'il fallait effectivement une réelle pluralité au sein de cette représentation même. Nous pouvons regretter toutefois qu'à l'occasion de cette nouvelle répartition des rôles, cette tendance ne prévoie pas la consultation consultation des populations, notamment sur les projets d'aménagement du quartier, pour lesquels elle devrait être systématique. Dans le monde entier, les villes deviennent ou redeviennent incontournables dans l'architecture territoriale des appareils publics

internationale. Grâce à sa gouvernance institutionnelle efficace et réactive et à son financement approprié, il doit permettre de s'adapter aux enjeux futurs et de faire rayonner les territoires environnants.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission, mes chers collègues, l'émergence du premier centre d'affaires européen, en l'espace de soixante ans, en lieu et place de pavillons vétustes voisins des bidonvilles et de petites usines de mécanique, ne s'est pas faite sans crise et sans rebond. Aujourd'hui, le quartier d'affaires de La Défense, vieillissant, cherche un nouveau souffle. C'est pour mieux penser l'avenir de La Défense, sa croissance comme le renouvellement de ses infrastructures, que le précédent gouvernement a souhaité réformer son schéma institutionnel. Il a voulu le faire tout d'abord en créant un établissement public unique, alors que jusqu'à présent aménagement et gestion du patrimoine étaient pensés au sein de deux entités distinctes. La cohérence des actions menées ne pourra qu'en être renforcée. Le précédent exécutif a également souhaité redonner la main aux principaux acteurs de ce territoire, les élus locaux. Il s'agit là d'une véritable révolution culturelle puisque, jusqu'à présent, la voix de l'État était prépondérante lorsqu'il fallait présider aux destinées du quartier d'affaires. Une prépondérance parfois toute relative, quand on sait combien les Hauts-de-Seine ont offert à la République d'illustres serviteurs de l'État. Le département des Hauts-de-Seine et sa majorité ont ainsi souvent pu trouver une oreille attentive auprès de l'État. Désormais les élus locaux vont acquérir une véritable liberté de gestion. C'est une revendication ancienne de la gauche dans ce département, et je m'en félicite, mais ces droits nouveaux appellent naturellement de nouvelles responsabilités. Durant plusieurs décennies, les collectivités situées sur le territoire de La Défense ont pu bénéficier de ressources très importantes sans nécessairement prendre part à l'entretien et à la réhabilitation du secteur. Ces ressources demeurent. Il y a une quinzaine de jours, la commune de Courbevoie a perçu 10 millions d'euros de droits de mutation liés à la vente de trois nouvelles tours de bureaux. Le 29 mars dernier, le conseil municipal de la ville de Puteaux a voté un budget de 430 millions d'euros, dont plus de 180 millions d'euros en investissement et près de 250 millions d'euros en fonctionnement. Pour mémoire, cette commune ne compte « que » 45 000 habitants. Il a donc été décidé d'instaurer un pacte de gouvernance engageant les collectivités concernées à abonder les ressources du nouvel établissement public à hauteur des besoins non couverts en matière de gestion, d'entretien et de remise en état du site. La rénovation du patrimoine de La Défense, dont l'urgence devient pressante, est estimée à un demi-milliard d'euros, peut-être plus. Cette régénération sera donc désormais essentiellement portée par par celles et ceux qui sont les premiers bénéficiaires de la richesse générée par ce site fort de 150 000 emplois et de plus de 3 millions de mètres carrés de bureaux. Cette remise à niveau viendra conforter les occupants actuels tout en permettant de saisir plus aisément les opportunités futures. Certes, la décision britannique de retrait des institutions européennes offre à la place de Paris et à son principal quartier d'affaires une attractivité nouvelle. Mais cette attractivité passera également par une évolution de son modèle de développement, trop monofonctionnel. Lors de la précédente législature, des efforts ont été menés pour humaniser et diversifier le quartier d'affaires. Ils devront se poursuivre. En conclusion, je veux saluer l'accord global qui a conduit à cette réforme. Il fait honneur au précédent gouvernement, qui a su une nouvelle fois démontrer son attachement à la décentralisation et à la mise en responsabilité de nos collectivités territoriales. C'est pour respecter l'équilibre de cet accord global que j'estime qu'il est nécessaire d'attendre la refonte de l'organisation du Grand Paris, annoncée par le Président de la République, pour réenvisager, au sein de ce nouveau schéma institutionnel, le rôle alloué à la métropole, aujourd'hui dotée de moyens bien trop modestes. Mais il ne faudra pas dans l'avenir occulter ce débat, car la vision métropolitaine est la plus à même d'oeuvrer efficacement au rééquilibrage des richesses créées au sein de la zone dense parisienne, qui demeure une terre de contrastes et de profonds

écoutés avec intérêt. Le précédent gouvernement a décidé le 10 mai de déposer ce texte, qui est, je l'ai dit tout à l'heure, le fruit de très longues discussions.

! Les modifications qui ont été apportées en commission suppriment de fait toute référence au périmètre d'intervention géographique de La Défense, ce qui ne nous paraît pas une bonne chose.

le cadre défini initialement par la loi d'habilitation qui organise la substitution des deux établissements dont c'est le périmètre actuel. Cet amendement vise par ailleurs à reprendre la proposition du Parlement de concentrer les communes sur le périmètre, tout en maintenant la procédure d'avis simple figurant au texte du Gouvernement. L'adoption de cet amendement nous permettrait donc de revenir à la cohérence et aux équilibres initiaux.

avec les méthodes qui sont les miennes, ce que je pense de ces modes de fonctionnement : comptez sur moi ! Quant aux responsables, je leur parlerai directement. Très

Il est d'usage que les établissements publics d'aménagement soient des outils pluriels, fédératifs, réunissant toutes les sensibilités politiques pour définir et construire des projets communs d'intérêt général.

À nos yeux, il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de désigner ses représentants au sein du conseil d'administration

comme si les 180 000 personnes qui y travaillent tous les jours n'avaient pas besoin de crèches pour leurs enfants, comme si les 45 000 étudiants de La Défense n'avaient pas besoin des différents services propres à la vie étudiante, comme si les 25 000 personnes qui habitent le quartier n'avaient rien à attendre en matière de vie quotidienne. Enfin, mes chers collègues, assurer le « bon fonctionnement des services publics », c'est aussi garantir la sécurité quotidienne. Comment ignorer cet aspect des choses à l'heure où les risques terroristes sont aussi importants ?

de suspendre le caractère exécutoire d'une décision de l'établissement qui irait à l'encontre du bon fonctionnement des services publics. Cette disposition était de veiller à la cohérence des opérations d'aménagement menées par les différents acteurs publics, qu'il s'agisse de l'établissement public, de l'État ou des pouvoirs locaux, dans un Grand Paris au développement rapide et complexe. Il est, certes,

puisse suspendre le caractère exécutoire d'une décision qui irait à l'encontre du bon fonctionnement des services publics. Il s'agit non pas de bloquer le fonctionnement du nouvel établissement,

du pouvoir du préfet, ce qui va bien au-delà des services publics. Dire que le préfet ne peut intervenir que sur les services publics, alors qu'il n'a pas à le faire

l'harmonie entre les différentes collectivités n'avait peut-être pas atteint un degré d'affection

il existe des risques de non-concordance entre des projets d'aménagement soutenu par l'établissement et des opérations nécessaires au bon fonctionnement des services publics- la RATP, SNCF Réseau, la SNCF ou la

commission, laquelle avait pour objet de simplifier la rédaction de l'ordonnance en prévoyant son entrée en vigueur au 1 janvier 2018, sans faire référence à la création de l'établissement public. Or l'article 34 de la constitution dispose clairement que la création d'un nouveau type d'établissement public relève du domaine de la loi. C'est la raison pour laquelle il nous paraît indispensable de mentionner dans l'ordonnance la date de création effective de l'établissement, en faisant référence à celui-ci. L'objet du présent amendement est donc de rétablir la rédaction initiale de l'ordonnance, pour des raisons juridiques.

La Défense compte aujourd'hui un peu moins d'une vingtaine de parcs de stationnement pour quelque 22 000 places de parking au total. Cela représente une manne financière, qui, chaque année, se compte en centaines de millions d'euros. On comprend donc que certains souhaitent l'accaparer, mais on peut douter que cela se fasse au nom de l'intérêt général. En restant propriétaire, avec une gestion confiée au nouvel établissement pour une durée de soixante ans, l'État aura la capacité d'attribuer les autorisations pour les cessions de places de stationnement. Cela signifie qu'il gardera un pied dans l'aménagement de La Défense, ce qui semble indispensable au vu des enjeux. Je tiens à préciser, en outre, que les salariés

issue des travaux de la commission, l'article 7 prévoit le transfert en pleine propriété des parcs de stationnement figurant dans le patrimoine de l'EPADESA. Le Gouvernement considère qu'il n'existe pas de motif d'intérêt général justifiant un transfert à titre gratuit des espaces de stationnement. Je vais vous démontrer

les revenus issus des parcs de stationnement sont attribués à celui-ci. C'est pourquoi le Gouvernement propose par cet amendement d'exclure les parcs de stationnement du transfert en pleine propriété des biens de l'EPADESA vers le nouvel établissement public Paris La Défense

Ces deux amendements de suppression soulignent l'imbroglio administratif et juridique qui entoure le quartier d'affaires de La Défense. La question cruciale est : qui est aujourd'hui propriétaire des parcs de stationnement ? L'EPADESA, l'un des deux établissements support du futur Paris La Défense, estime qu'ils sont à lui. L'article 55 de la loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, dont j'étais rapporteur, prévoit dans ses dispositions d'habilitation une substitution du nouvel établissement aux deux anciens, dans leurs droits et obligations, donc en matière de parcs de stationnement. Eh oui quant à lui, que les parcs lui appartiennent et que rien ne justifie un tel transfert. On peut regretter l'absence de réponse du préfet de région à mes sollicitations pour recueillir son avis sur l'ordonnance, et surtout l'exposé des motifs très

ne justifie l'absence de transfert des parcs de stationnement, sauf à vouloir complexifier la gestion de ce quartier. Or cette complexité est précisément à l'origine de notre débat aujourd'hui, vous l'avez

que j'ai menées, on m'a signalé des dossiers dignes de Gabriel Chevallier, dont certains ont dû être tranchés par le Premier ministre lui-même. En refusant le transfert des parcs de stationnement, on ne ferait que laisser perdurer une situation dénoncée

je ne comprends même pas que l'on se pose la question

J'ai même proposé de sous-amender l'amendement du Gouvernement ! Je déplore le refus qui m'a été opposé. Je considère que l'esprit de l'article

pour les communes concernées. La ville de Nanterre serait dépossédée des ZAC des Groues et de Seine Arche, des quartiers d'habitation qui comprennent notamment des services publics et des établissements scolaires,

Violant le principe constitutionnel de libre administration des collectivités et de non-tutelle d'une collectivité sur l'autre, on mettrait une ville de 93 000 habitants devant le fait accompli, sans aucune consultation. jamais, j'insiste ! -la ville de Nanterre, principale concernée, n'a donné son accord sur un tel projet. Bien au contraire ! Le maire de Nanterre, auditionné par

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.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

n° 124 : Le Sénat a adopté. La commission de la culture a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires. La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement. En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame M. Jean-Pierre Leleux membre titulaire et Mme Françoise Férat membre suppléant de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, ainsi que M. Christian Manable membre de la Commission supérieure